du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010 837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Que se passe t il ? Y aurait il du gaz dans l’hydrogène vert ? Alors qu’il est urgent de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles russes et d’accélérer la transition écologique, la formidable ambition de réduire les émissions de CO2 des aciéries n’a de sens que si elle repose sur la production d’hydrogène issue d’énergies renouvelables décarbonées à bas coût, laquelle favoriserait le développement d’une filière industrielle prometteuse autour de l’éolien offshore et de l’électrolyse dans les ports verts de la Méditerranée, comme Fos sur Mer et Port la Nouvelle.

ci s’engagent à diviser par deux leurs émissions de gaz à effet de serre en dix ans. Le 26 novembre 2023, chacun de ces sites a signé avec l’État

doté de 4 milliards d’euros, une somme prise sur l’enveloppe budgétaire de la stratégie nationale hydrogène. À ce mécanisme s’ajoutera un soutien à l’adaptation des procédés industriels, financé par l’enveloppe budgétaire consacrée à la décarbonation de l’industrie, qui permettra de maintenir l’excellence technologique française en matière de sidérurgie. Ces deux dispositifs, qui pourront profiter aussi bien aux industriels historiques qu’aux start up innovantes, assureront la pérennité de la production d’acier décarboné sur le site de Fos sur Mer. La parole

pour rendre cette mutualisation plus contraignante, dès lors que cela est possible et n’affecte pas la qualité du réseau ? La parole est à Mme la ministre

une solution. Les entreprises relevant du registre du commerce et des sociétés ont ainsi la possibilité d’utiliser Infogreffe à titre dérogatoire depuis le guichet unique, et d’obtenir ainsi un extrait Kbis actualisé. Pour les autres entreprises, le recours à des formulaires papier est possible dans certains cas exceptionnels. Les fonctionnalités et l’ergonomie du guichet et du registre national des entreprises progressent en tenant compte des avis des organismes destinataires des formalités, dont font partie les avocats, ainsi que de ceux de panels d’entreprises et de professionnels des formalités.

d’achat de ces salariés vient s’ajouter à plusieurs réorganisations n’ayant qu’un seul but : réduire les dépenses de personnel en exigeant toujours plus de polyvalence des travailleurs. Un pouvoir d’achat en baisse et une organisation du travail toujours plus stressante, c’est malheureusement le lot de millions de salariés dans notre pays aujourd’hui. Auchan, cette situation est encore aggravée par les profonds bouleversements qui perturbent la grande distribution, notamment en raison de la faillite du groupe Casino. Pour Auchan et ses salariés, les conséquences de cette situation sont majeures. Alors que le groupe enregistre un déficit de 379 millions d’euros, le rachat d’une centaine de magasins Casino va peser lourd.

». Enfin, pour les producteurs, le déséquilibre dans les négociations commerciales va encore s’accentuer. Avec ce mouvement de concentration des acteurs, les géants de la distribution vont en effet y gagner dans le rapport de force actuel, et pas seulement face aux grandes multinationales de l’agroalimentaire. Pour les petits producteurs, ce sera plus que jamais le pot de terre contre le pot de fer en matière de fixation des prix et de qualité des produits. Après ces deux journées de mobilisation à Auchan, quel rôle le Gouvernement entend il jouer pour que les salariés ne soient pas les grands perdants de la politique du groupe ? Sur un plan plus prospectif, comment le Gouvernement compte t il prévenir les conséquences des grandes manœuvres engagées dans le secteur de la distribution à la suite de l’effondrement du groupe Casino pour les salariés, les consommateurs et les fournisseurs ? La parole est à Mme la ministre

afin que celui ci ait le temps de trouver la meilleure solution pour résoudre ses difficultés. Cet effort exceptionnel a permis la conclusion, sous l’égide de l’État, d’un accord global solide, qui devrait assurer la pérennité du groupe, et en particulier de ses commerces de proximité et de la plupart de ses 50 000 emplois en France. Cependant, la très forte dégradation de l’activité du groupe l’a contraint à céder ses hypermarchés et supermarchés à Auchan et au Groupement Les Mousquetaires. Cette solution, qui repose sur deux acteurs de premier plan de la grande distribution française, offre des perspectives à la quasi totalité des hypermarchés et supermarchés et à l’ensemble de leurs salariés.

l’adoption de loi relative à l’énergie et au climat, qui est venue concrétiser la promesse du Président de la République d’arrêter définitivement ce mode de production d’électricité en 2022, ce choix s’est révélé visionnaire. Si différents facteurs, dont la guerre en Ukraine, expliquent le retard pris dans la fermeture des centrales à charbon, le Président

en centrales à biomasse. Or la direction d’EDF, entreprise pourtant détenue par l’État français, prend le contrepied de ces annonces présidentielles. En effet,

que les hypothèses les plus pessimistes. Le prix de l’électricité ainsi produite serait alors prohibitif… Il est inacceptable qu’une entreprise nationale agisse à l’encontre de politiques décidées au plus haut niveau de l’État, surtout lorsque celles ci concernent la sécurité de l’approvisionnement électrique de nos territoires.

Sa fermeture, initialement prévue le 1 janvier 2022, a été repoussée de manière à garantir la sécurité d’approvisionnement électrique face aux difficultés rencontrées durant les hivers 2022 et 2023. Le Président de la République s’est effectivement engagé à ce que la France sorte définitivement du charbon d’ici le 1 janvier 2027. Cet engagement s’inscrit dans l’ambition globale du Gouvernement de faire de la France la première grande nation verte à sortir des énergies fossiles.

Le projet a finalement été abandonné par les deux acteurs, faute d’un modèle économique satisfaisant et d’un retour d’expérience suffisant sur la technologie envisagée. Les discussions ont néanmoins repris autour d’un projet Ecocombust 2

disposition législative qui a interdit la réduction du débit d’eau résulte en fait d’une maladresse rédactionnelle, comme on peut le constater à la lecture des débats parlementaires de l’époque. Toujours est il que la réglementation actuelle pénalise les distributeurs, qui estiment être démunis de tout moyen d’action face aux impayés. Ils décident par conséquent d’arrêter le financement des travaux inscrits aux plans pluriannuels d’investissement et craignent parfois – c’est le cas en Isère

du code de l’action sociale et des familles, a interdit les coupures d’eau pour impayés à toute époque de l’année pour l’ensemble des résidences principales, sans condition de ressources. Pour autant, l’interdiction des coupures d’eau n’emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l’abonné. Le Gouvernement est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer dans la gestion du service public de l’eau potable. Cet état du droit pourrait encourager les comportements inciviques et avoir des effets financiers notables, non seulement pour les services, en raison

pour adresser au débiteur une mise en demeure ou lui signifier une sommation de payer. Il est également possible de mettre en place une solution de paiement échelonné après étude et analyse de la situation. Si les démarches amiables restent vaines, l’entreprise peut en outre engager une procédure judiciaire pour procéder au recouvrement, légitime, de sa créance. J’ajoute,

comme vous le savez, le choucas des tours est inscrit à l’annexe II de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages. Cette annexe énumère les espèces d’oiseaux pouvant être chassées dans certains États membres seulement. En cohérence avec les dispositions de cette directive, l’espèce est protégée en droit français et n’est donc pas chassable. Le statut de protection du choucas des tours permet néanmoins des destructions à titre dérogatoire,

Afin de limiter les dommages causés aux agriculteurs, la maîtrise des populations de choucas des tours doit par ailleurs impliquer, au delà des tirs létaux, une approche préventive, comprenant des dispositifs innovants de protection des cultures et d’effarouchement et la limitation de l’accès aux sources de nourriture, ainsi qu’aux sites de nidification comme les cheminées. Afin de mettre

Le premier comité de pilotage de ce plan s’est tenu en mars 2023 ; il a rassemblé l’ensemble des acteurs concernés des quatre départements bretons. Le second doit se tenir à la fin de ce mois d’avril 2024 ; il permettra de finaliser ce plan et d’en mettre en œuvre toutes les actions, au

De nombreux petits syndicats des eaux de mon département sont en grande difficulté. Je pense tout particulièrement au syndicat des eaux du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN), qui ne sait plus comment assumer ses charges d’investissement pour se conformer à une réglementation toujours plus stricte et pas toujours très lisible, entre les prescriptions de l’Agence nationale de dont la rigueur a été majorée par des captages d’eau dans des nappes très basses l’année dernière. Dans la conjoncture inflationniste que nous connaissons, les usagers et les collectivités ne sont plus en mesure d’absorber ces hausses tarifaires exorbitantes. Pourtant, suite de la transposition de la directive européenne sur l’eau potable, l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine prévoyait bien la compensation financière par l’État de l’accroissement des charges des collectivités résultant de ces nouvelles obligations. Or aucun crédit dédié n’a été inscrit dans la loi de finances pour 2024, qui engage cependant la réforme d’envergure des redevances des agences de l’eau et la refonte des redevances « petit cycle de l’eau », prévue pour le 1 janvier 2025.

qui n’ont plus la surface financière suffisante pour supporter seuls l’ensemble des coûts induits par la mise en conformité de leurs installations. La leurs installations. La parole est à M. le ministre délégué. Madame la sénatrice Pluchet, la contamination des ressources en eau destinées à la consommation humaine constitue une situation préoccupante pour de nombreuses collectivités responsables de la distribution de l’eau, notamment pour les syndicats des eaux du département de l’Eure. Je le rappelle, en cas de dépassement de la limite de qualité, les personnes responsables de la distribution d’eau doivent déposer une demande de dérogation qui, pour être validée, doit s’accompagner d’un plan d’action permettant le respect de la limite de qualité sous une période de dérogation ne pouvant pas excéder trois ans. Comme vous le savez, un appui aux investissements et à l’emprunt pour les collectivités concernées peut être apporté par la Banque des territoires l’octroi de prêts à moyen terme ou à long terme Ces prêts font partie intégrante du plan Eau, qui a été annoncé par le Président de la République au mois de mars 2023. Ils connaissent un réel succès depuis leur lancement. Afin de répondre à la demande des collectivités, l’enveloppe budgétaire qui leur est consacrée a été doublée : elle s’élève à 4 milliards d’euros pour la période 2023 2027. La Banque des territoires a également développé une offre d’accompagnement gratuite à destination des collectivités, nommée Aquagir. Celle ci porte sur toute la gestion du cycle de l’eau et comprend un volet relatif à la production d’eau potable.

qui accompagnent les collectivités, les industriels, les agriculteurs dans leurs projets d’investissement permettant de faire converger la transition écologique et le développement des territoires. Pour la deuxième année de la mise en œuvre du plan Eau, la priorité est donnée à la préservation de la qualité de l’eau. Le relèvement important du plafond de recettes des agences de l’eau prévu par la loi de finances pour 2024 vise justement à assurer le financement de certaines mesures destinées à renforcer la protection des aires d’alimentation de captage. C’est ainsi que, par l’intermédiaire des agences de l’eau et des interventions financières définies dans leurs programmes pluriannuels d’intervention, le soutien aux actions favorisant la reconquête de la qualité de l’eau, notamment les pratiques agricoles à bas niveau d’intrants, a été renforcé dans ces aires d’alimentation de captage.

Chaque déclaration comporte l’identité et l’adresse du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l’identité, l’adresse et le numéro d’agrément du ou des piégeurs, ainsi que le lieu dit du piégeage. Dans un avis de 2021, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a rappelé que ces documents étaient communicables à toute personne en faisant la demande. des maires décident volontairement de ne pas transmettre les listes de déclaration de piégeage des animaux classés nuisibles aux personnes qui les sollicitent. Ils se retrouvent de fait poursuivis en justice par ces dernières pour non communication. Si ces élus choisissent de se soustraire à une telle demande, c’est par crainte que certains individus ne s’en servent pour aller détruire les pièges mis en place ou bien encore pour effacer les marquages obligatoires sur ceux ci, afin de les rendre non conformes à la législation et d’appeler ensuite l’Office français Des exemples illustrent une telle manière de faire dans d’autres départements. Et, dans des cas plus extrêmes, certains vont jusqu’à menacer les piégeurs, voire ceux qui ont demandé la mise en place des pièges… Rappelons qu’il existe beaucoup d’individus désireux d’entraver la mission qu’accomplissent les piégeurs dans notre pays. Il est à craindre que beaucoup de ces derniers ne finissent par jeter l’éponge face aux attaques qu’ils subissent, alors même qu’ils sont un outil de régulation essentiel de la faune sauvage.

Comme vous le savez, l’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques est l’un des piliers de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France le 8 juillet 2002. Aussi, le principe établi dans la loi est celui d’une communication des documents administratifs pour des questions de transparence de l’action publique.

conformément à l’article L. 311 6 du code des relations entre le public et l’administration, il est prévu que ne sont pas communicables aux demandeurs les documents administratifs dont la communication « porterait atteinte à la protection de la de la vie privée ». De plus, les dispositions de l’article L. 311 5 du même code s’appliquent dans la mesure où elles précisent que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte » à la « sécurité des personnes ». Or les piégeurs, une fois identifiés et localisables, peuvent faire l’objet d’agissements visant à porter atteinte à leur intégrité physique ou morale, à leurs biens ou à la bonne réalisation de leur mission. Au vu des deux dispositions législatives que je viens de citer et du contexte de la demande, les maires comme les préfets peuvent répondre défavorablement ou partiellement à certaines requêtes. Une demande de modification de l’arrêté du 29 janvier 2007 définissant la liste de documents à fournir pour une déclaration de piégeage, et notamment de son article 11, a été évoquée lors de la dernière assemblée générale de l’Union nationale des associations de piégeurs

du futur dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR). À partir du 1 juillet, le programme FRR remplacera les zones de revitalisation rurale (ZRR). Il permet aux communes de proposer des exonérations fiscales aux professionnels qui s’y installent et s’accompagne de dotations supplémentaires pour celles ci. La communauté de communes du Réolais n’y est malheureusement pas éligible, car la densité de population est un peu au dessus du critère défini par la loi. Pourtant, elle coche tous les autres critères de précarité ! La fragilité sociale et économique du Réolais est reconnue par l’ensemble des institutions. Ce territoire fait en effet partie du « croissant de pauvreté de la Gironde », l’établissement public de l’indice de fragilité sociale de la ville de La Réole, déterminé par les services du département, s’établit à 1,5, soit le plus haut niveau possible. Enfin, le secteur est particulièrement déficitaire en offre de soins, alors que sa population est précaire et vieillissante : chaque médecin y prend en charge environ 1 460 patients, et 2 500 habitants sont encore sans médecin traitant. De plus, toutes les communautés de communes autour du Réolais sont classées en zone de revitalisation rurale et bénéficieront du futur dispositif FRR à la faveur d’une densité plus faible, ce qui risque d’induire une concurrence déloyale entre les collectivités de communes limitrophes.

pour soutenir la population de la communauté de communes du Réolais et s’il serait possible d’assouplir le dispositif pour que les communautés de communes avec des populations particulièrement précaires et dont toutes les communes limitrophes bénéficient du dispositif FRR

les territoires. La parole est à M. le ministre délégué. Madame la sénatrice Lassarade, les zones de revitalisation rurale arrivaient à échéance au 31 décembre 2023. Il était donc indispensable de les réformer, afin que les territoires ruraux puissent continuer à bénéficier du soutien dont ils ont besoin. Inchangées depuis 2015, zonant 13 400 communes sur critère et ayant maintenu artificiellement 4 000 communes alors qu’elles ne répondaient plus aux critères de zonage, les ZRR étaient devenues injustes injustes et inéquitables. Après un an et demi de consultation, la réforme des ZRR, devenues le dispositif France Ruralités Revitalisation, a été adoptée à l’unanimité dans votre hémicycle lors de l’examen de la loi de finances pour 2024. C’est une réforme généreuse, qui zone désormais de droit 17 700 communes en tenant compte au maximum des spécificités des territoires de montagne ou des départements très peu densément peuplés. Pour ce qui est de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, composée de 41 communes, 11 communes avaient été maintenues artificiellement dans le zonage en 2015, puisqu’elles ne répondaient déjà plus aux critères, et 30 n’étaient pas zonées. En effet, avec la réforme FRR, ces 11 communes ne sont plus zonées. Comme tout zonage, il y a des entrants et des sortants. Sur les 2 200 communes sortantes, 1 802 ne répondaient déjà plus aux critères de zonage en 2015 ; cela représente 81,9 % des communes sortantes. Dominique Faure étudie en ce moment des alternatives pour lisser au maximum les effets de seuil et accompagner au mieux ces communes. communes. Les communes de la communauté de communes du Réolais, dont la densité est de 73,5 habitants par kilomètre carré, demeurent très éloignées du seuil, fixé à la médiane, c’est à dire à 63,57 habitants par kilomètre carré. Cependant, madame la sénatrice, nous sommes conscients

en 2026, la loi prévoit que les communautés de communes pourront déléguer par convention tout ou partie de ces compétences à leurs communes membres, ainsi qu’à leurs syndicats existants au 1 janvier 2019 2019 et dont le périmètre est infracommunautaire. Dans ce cas, les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte des communautés délégantes. Cette possibilité est le principal assouplissement apporté au transfert obligatoire de ces deux compétences en 2026. Les communautés de communes sont confrontées à différentes interrogations. D’abord, dans le cadre de la gestion déléguée, elles souhaitent savoir s’il peut y avoir des tarifs différents pour chaque commune ou syndicat délégataire et, le cas échéant, si ces tarifs doivent être fixés par la communauté de communes ou par les délégataires communaux ou syndicaux. Ensuite, elles demandent si les budgets annexes dont disposent actuellement les communautés ou leurs syndicats pour ces compétences doivent être transférés aux communautés de communes en l’état ou clôturés concomitamment au transfert de compétences. Dans tous les cas, elles s’interrogent sur le sort qui sera réservé dans une telle situation au au solde des budgets annexes communaux, aux syndicats préexistants, au transfert et à la gestion déléguée. Enfin, dans le cas d’une gestion déléguée, elles demandent si chaque commune ou syndicat délégataire doit disposer d’un budget annexe rattaché à son budget principal pour l’eau et l’assainissement ou s’il appartient au contraire aux communautés délégantes de disposer d’autant de budgets annexes que de délégataires sous sa responsabilité. Ces questions sont importantes. D’ailleurs, il serait peut être bon qu’un

Toutefois, ce transfert ne signifie pas une harmonisation immédiate des tarifs. Les différenciations tarifaires pourront exister sur le territoire communautaire du fait du maintien des tarifs précédemment fixés par les communes. Comme le préconise une instruction du 18 septembre 2017, l’harmonisation tarifaire devra intervenir dans un délai raisonnable. Ainsi, des différences tarifaires au sein de la communauté de communes ne sauraient perdurer définitivement, sauf à méconnaître le principe d’égalité, auquel il ne peut être dérogé que dans des limites fixées de longue date et de manière constante par la jurisprudence. S’agissant de l’exercice des compétences eau et assainissement, la communauté de communes peut choisir de déléguer tout ou partie de ses compétences à une commune membre ou à un syndicat infracommunautaire. Dans ce cas, les compétences sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. Ainsi, la délégation ne peut pas faire obstacle au principe d’égalité de traitement des usagers service. Pour les communautés de communes, il est nécessaire de mettre en place un budget annexe unique par compétence, c’est à dire un budget annexe pour la compétence eau et un budget annexe pour la compétence assainissement, quel que soit le nombre de délégations existantes. Pour les communes, il est préconisé de créer un budget annexe dédié à chaque compétence déléguée. Pour les syndicats, le maintien des budgets annexes

qui incite notamment à réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation. La population de chats est estimée à plus de 13 millions, et un couple de chat peut donner naissance à 20 000 petits en quatre Bien que la stérilisation ne soit toujours pas obligatoire, c’est bien la seule action efficace pour endiguer la prolifération des félins laissés en liberté. Les maires sont, une fois encore, en première ligne, aidés par l’article L. 211 27 du code rural et de la pêche maritime, qui leur permet de faire procéder à la capture des chats errants, en vue de les stériliser et identifier, puis de les relâcher. Mais, devant l’ampleur croissante du phénomène et les coûts d’intervention, nous avons introduit dans la loi de finances pour 2024 une dotation exceptionnelle pour la stérilisation des chats. Or, malheureusement, à l’heure actuelle, aucune directive n’a été communiquée concernant la procédure pour bénéficier de cette dotation. Le Gouvernement peut il nous communiquer les modalités, ainsi que les conditions d’accès à cette aide financière pour les communes qui désirent en bénéficier ? La parole est

parole est à M. le ministre délégué. Monsieur le sénateur Hugonet, vous m’interrogez sur les modalités d’accès à la dotation exceptionnelle de 3 millions d’euros pour la stérilisation des chats, adoptée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2024, sur une initiative parlementaire. Ces nouveaux crédits, introduits par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, ont vocation à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place d’une stérilisation efficace des chats sauvages.

C’est la raison pour laquelle un décret de transfert de crédits entre les programmes budgétaires des deux ministères est prévu. Ce transfert interviendra, à l’instar de l’ensemble des décrets de transfert, avant la fin du premier semestre 2024. Les modalités et les conditions d’accès à cette aide financière seront donc précisées à cette même occasion

De nombreuses collectivités, notamment rurales, sont propriétaires de bâtiments anciens transformés en logements et loués à des prix attractifs, permettant l’installation de nouveaux habitants dans ces communes, où l’offre de location est bien souvent saturée ou inexistante.

qui risquent de peser lourd dans les budgets communaux. Il apparaît donc tout à fait essentiel que l’État accompagne financièrement les collectivités pour permettre d’atteindre cet objectif national, d’autant que les règlements de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) excluent la plupart du temps

MaPrimeRénov’ est une aide publique destinée à financer les travaux pour améliorer la performance énergétique des logements du parc privé. Elle est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements de ce parc pour les logements qui sont construits depuis au moins quinze ans, occupés à titre de résidence principale, que le propriétaire occupe les lieux ou en fasse bénéficier un locataire. À ce stade, il n’est pas prévu de l’élargir au parc social ni aux logements détenus par les personnes publiques. Il existe néanmoins d’autres financements pour soutenir la rénovation énergétique des logements que vous évoquez dans votre question. Ainsi, depuis 2023, une mesure spécifique est dédiée dans le fonds vert pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur projet de rénovation énergétique. Elle vise tous les bâtiments des collectivités, y compris les bâtiments avec logements, et soutient les projets de rénovation permettant d’atteindre une baisse des consommations d’énergie d’au moins 40 %. Les logements communaux sont ainsi éligibles à la mesure de rénovation énergétique des bâtiments locaux du fonds vert. Pour autant, ce dernier n’ayant pas vocation à se substituer à d’autres financements, il convient de mobiliser en priorité les subventions publiques dédiées à la rénovation des logements, en particulier le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) pour les logements conventionnés à l’aide personnalisée des collectivités. Le sujet de l’habitat est également présent au cœur du plan France Ruralités, sur lequel Mme Dominique Faure s’est engagée pour sortir des logements de la vacance. Vous savez que notre pays compte un taux de logements vacants de plus de 8 % ; c’est significatif.

en partance et en provenance de l’aéroport d’Orly. Notre compagnie, pourtant nationale, ne desservira donc plus Nice, Marseille ou encore Toulouse dès 2026. Il s’agit d’une décision brutale, lourde de conséquences, prise sans aucune concertation avec les élus et acteurs concernés ! Ce sont pourtant ces derniers qui, par leur travail de qualité, permettent d’attirer les voyageurs vers nos territoires, et ce grâce à des événements de renommée mondiale. Sénatrice des Alpes Maritimes, mais aussi présidente du comité régional du tourisme Côte d’Azur France, je le regrette sur un plan non seulement humain, mais également économique, puisque nous sommes la première destination touristique après Paris. Cette dégradation de l’offre et à juste titre ! J’ai saisi le Gouvernement. Avec Éric Ciotti, nous avons rencontré les syndicats du personnel, très inquiets, comme vous vous en doutez. Puis, nous avons alerté – encore ! – le Premier ministre, le 2 avril dernier, afin que la compagnie prenne le temps de la concertation. Je le précise, l’alternative ferroviaire n’est pas une option crédible pour nous. Un trajet en train entre Nice et Paris, c’est, en moyenne, sept heures : un déplacement pour un rendez vous professionnel dans la journée est donc impossible ! Vous allez me répondre que le Gouvernement sera « attentif » à la situation. Mais le président de Transavia a refusé de s’engager à maintenir les créneaux actuels d’Air France et la qualité du service sera inférieure

publiquement regretté cette décision et s’est engagé à mener une concertation avec les élus. Quatre mois plus tard, toujours rien ! Je vous le demande solennellement : quand serons nous associés au devenir des liaisons opérées par la filiale d’Air France entre Paris et nos territoires ? La parole est à M. le ministre

Durant cette crise, les organisations et les habitudes de travail ont – vous le savez – profondément évolué et entraîné une baisse du trafic aérien lié au voyage d’affaires, en particulier sur les liaisons de et vers Paris. Alors que, dès novembre 2023, le trafic aérien en France a retrouvé son niveau de 2019, la fréquentation sur les lignes radiales du trafic domestique dépassait à peine 70 % de son niveau d’avant crise au mois de février. Le trafic de la navette Orly Nice a baissé de près de 60 par rapport à 2019. La clientèle d’affaires est ainsi passée d’un peu plus de 100 000 passagers en 2019 à 50 000 en 2023. Dans ce contexte, il est souhaitable qu’Air France mette en œuvre des solutions permettant d’améliorer sa rentabilité ; c’est la condition de sa pérennité face à la concurrence. Toutefois, le Gouvernement vous rejoint sur le fait que ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des territoires et de leur connectivité. Le groupe a bien confirmé que cette évolution s’accompagne, d’une part, du renforcement des liaisons opérées par Air France de Nice vers Paris Charles de Gaulle, dont le nombre de rotations est passé de sept par jour en 2019 à dix par jour à l’été 2024 et continuera d’augmenter, et, d’autre part, du développement des liaisons de Transavia vers Paris Orly. La compagnie Transavia, en pleine croissance, pourra utiliser sur ses lignes au départ d’Orly les nouveaux Airbus A320neo, qui remplacent progressivement depuis 2024 les Boeing 737 d’ancienne génération, ce qui est – nous le pensons – un gage d’amélioration des conditions de transport des passagers. Le Gouvernement est conscient de l’importance du maintien de la connectivité de Nice et de la Côte d’Azur.

contre les fantassins de la République. Et malgré les discours de fermeté, la situation ne cesse de se dégrader ! Le Sénat a pris ses responsabilités en adoptant un texte fort, que j’ai soutenu, et en trouvant un accord avec nos collègues de l’Assemblée nationale, le 27 février dernier. vise un double objectif : d’une part, mieux protéger les élus locaux dans l’exercice de leur mandat et, d’autre part, améliorer l’accompagnement par les acteurs judiciaires et étatiques chargés des élus victimes. Toutefois, renforcer notre arsenal législatif ne peut pas être l’unique réponse à ce fléau qui s’enracine. Le mal est profond, c’est celui de la perte de l’autorité de l’État. Or, sans une extrême fermeté envers ceux qui font désormais de la violence un mode d’expression comme un autre, nous n’y arriverons pas. Monsieur le ministre, la tolérance zéro doit être la règle, sans excuses ni faux fuyants. Le sentiment d’impunité doit être combattu sans faiblesse, et la loi doit être appliquée réellement. La protection des élus contre les agressions est une condition du respect de l’État de droit. Aujourd’hui, plus que jamais, compte tenu des fractures de la société française, les élus locaux sont le ciment de la vie démocratique de notre pays. Monsieur le ministre délégué, au delà de l’indignation, entendrez vous le cri d’alarme, voire de détresse qu’ils vous adressent

Dire cela est une évidence, mais le rappeler est une nécessité et un devoir. Je vous remercie donc de votre question, qui me permet de faire un point d’étape sur le sujet au nom du Gouvernement.

: c’est heureux, et nous pouvons collectivement nous en féliciter. Comment répondons nous concrètement à ces violences ? Tout d’abord, le réseau de référents élus au sein des forces de l’ordre est désormais structuré et connu, coordonné par le centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, spécialement créé pour l’occasion. Plus d’un million d’euros ont déjà été engagés pour équiper nos forces de sécurité intérieures de caméras judiciaires pour la protection ponctuelle des domiciles des élus menacés. Par ailleurs, 2,5 millions d’euros seront très prochainement débloqués pour garantir la protection physique des élus locaux. Des boutons d’appel discrets sont actuellement déployés dans chaque préfecture en vue d’être prêtés aux élus faisant l’objet de menaces particulièrement graves. Enfin, depuis novembre dernier, une ligne de soutien psychologique est consacrée aux élus,

certains territoires dans le Morbihan sont soumis à une tension foncière et immobilière qui s’accroît en proportion de leur attractivité résidentielle, touristique et patrimoniale. Les actifs locaux n’ont plus accès à une offre résidentielle abordable, ce qui entraîne des difficultés de recrutement dans les différents métiers exercés

Détenus par les organismes de foncier solidaire (OFS), les terrains peuvent ensuite être loués, un bail emphytéotique d’une durée comprise entre 18 et 99 ans.

visent les mêmes objectifs d’accession aidée, ciblent le même public, bénéficient de la même fiscalité – une TVA à 5,5 % – et constituent un outil de maîtrise de la production de logements

Ce dispositif purement administratif, sans conséquence économique pour les finances publiques – si ce n’est un meilleur contrôle du niveau de fiscalité réduite accordé –, permettrait à la collectivité de maîtriser sa politique publique de l’habitat en fonction de la réalité des besoins de son territoire. Outre le fait que ces logements ne sont comptabilisés qu’à la livraison dans le bilan triennal, contrairement aux autres logements qui sont comptabilisés à la délivrance de l’agrément, cela permettrait à un territoire de ne pas se laisser déborder par une production excessive

consent à un preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession sociale à la propriété de logements, sous conditions de ressources. Seuls les organismes de foncier solidaire, qui sont des organismes à but non lucratif ou à lucrativité limitée – le plus souvent des bailleurs sociaux et qui ont été agréés par le préfet de région, sont autorisés à conclure un BRS. L’agrément d’un OFS est accordé après instruction par les services de l’État et avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), dont un des collèges est composé de représentants des collectivités. À ce titre, les services de l’État et le CRHH analysent le programme prévisionnel des actions de l’organisme concerné et des modalités de contrôle de l’affectation des baux qu’il entend pratiquer, principalement dans les zones tendues ou très tendues. Cette procédure d’agrément sera par ailleurs renforcée réglementairement, afin que le préfet puisse examiner plus précisément l’adéquation de la cible du futur OFS avec les politiques locales de l’habitat définies notamment dans le Ainsi, un organisme demandant l’agrément OFS devra désormais présenter une étude de marché justifiant la manière dont il entend répondre au besoin spécifique de logements en accession sociale sur le territoire concerné et pour la population qui y réside. Chaque vente en BRS fait également l’objet d’une analyse par l’OFS lui même. L’organisme vérifie que le ménage correspond à la population cible du BRS en contrôlant notamment la situation fiscale de ce dernier et le respect des conditions de ressources. L’adéquation entre l’activité de l’OFS et la réponse aux besoins en matière d’accession sociale à la propriété sur le territoire concerné est enfin contrôlée annuellement par l’État. En effet, chaque OFS a l’obligation de transmettre, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, un rapport d’activité au préfet. Dans ce rapport, l’OFS doit transmettre la liste des bénéficiaires de baux réels solidaires, ainsi qu’un bilan du suivi de la situation de ces bénéficiaires

ne dispose sur son territoire que de 13 % de logements sociaux au lieu des 20 % exigés par la loi. Cette appréciation occulte la réalité des efforts que cette commune, comme tant d’autres, consacre à se conformer à la loi.

Sanctionner par de lourds prélèvements pécuniaires des communes qui emploient par ailleurs des centaines de milliers d’euros et, donc, une large part de leurs ressources à des aménagements préparatoires indispensables à l’accueil de nouveaux logements sociaux – voirie, acquisition de terrains – est une injure faite à la bonne volonté de ces maires. En effet, sauf à abdiquer tout bon sens et à urbaniser leurs communes de façon anarchique, les édiles ne peuvent atteindre cet objectif que de manière progressive et linéaire. Cela suppose donc de leur laisser le temps d’inscrire cet objectif dans une trajectoire pluriannuelle. On ne saurait attendre d’eux qu’ils fassent sortir de terre des centaines de logements sociaux d’une année sur l’autre. Il serait plus conforme à l’esprit de la loi SRU d’apprécier les efforts des communes,

à l’heure où l’injonction à la mixité sociale se conjugue avec celle de la sobriété foncière et alors que les ressources financières des collectivités sont plus contraintes que jamais – la situation pourrait d’ailleurs empirer –, laisserez vous cette aberration se perpétuer ?

plusieurs mécanismes permettent déjà d’adapter le dispositif SRU aux particularités des communes concernées, en particulier les plus petites. Le législateur a d’ailleurs renforcé cette logique de différenciation à la faveur de la loi du Ainsi, le prélèvement supporté annuellement par les communes déficitaires, qui est proportionnel à leur déficit en logements sociaux et à leur potentiel fiscal, est adapté à leur situation et aux efforts qu’elles déploient. En ce sens, des exonérations de prélèvements sont prévues, notamment pour les 10 000 communes bénéficiant de la part cible de la dotation de solidarité rurale (DSR), sous réserve que celles ci disposent d’une part minimale de logements sociaux. En outre et surtout, les communes peuvent diminuer leur prélèvement à hauteur des dépenses qu’elles ont engagées pour la production de logements sociaux, comme le financement d’études ou leurs efforts pour minorer le coût Dans tous les cas, il est essentiel de rappeler que ce prélèvement ne constitue en aucun cas une pénalité. Les sommes prélevées sont versées à l’intercommunalité délégataire des aides à la pierre et réservées à la construction de logements sociaux. Le prélèvement SRU est ainsi l’un des moteurs de la production de logements sociaux dans le pays. Si toutefois une commune rencontre des difficultés objectives à respecter ses obligations et ne peut être exemptée, elle peut toujours signer un contrat de mixité sociale lui permettant, si sa situation le justifie,

qu’elle soit d’origine renouvelable ou non renouvelable. Toutefois, ce dispositif Éco énergie tertiaire n’impose pas que l’installation photovoltaïque sur le toit des bâtiments soit financée par son propriétaire. L’origine renouvelable de l’énergie – ici de l’électricité – ne doit pas être considérée comme un droit à consommer davantage. Si la production d’énergie renouvelable est vertueuse, il convient d’être vigilant sur l’impact des installations de production sur l’environnement lorsqu’aucun effort n’est fait pour réduire la consommation. La pose

cadre des appels d’offres lancés régulièrement par le ministère. Ces collectivités peuvent également bénéficier d’une prime à l’autoconsommation si le développement du photovoltaïque s’inscrit dans une logique de réponse à un besoin de consommation

des armées. Notre calendrier annuel est rythmé par les cérémonies patriotiques permettant de commémorer les anciens combattants. Les porte drapeaux ont une mission hautement symbolique, puisqu’ils rendent hommage aux combattants et disparus en portant le drapeau tricolore de leur association. L’importance mémorielle et symbolique donnée à cette tradition française du souvenir ne trouve cependant aucun financement public d’importance équivalente. Très bien imposée par un certain code vestimentaire, les accessoires et le matériel pour les cérémonies ne sont pas toujours subventionnés par les collectivités, ou le sont de manière insuffisante.

la bienvenue. Alors que le Président de la République veut mettre l’accent sur la formation des jeunes, sur ce qui fait notre histoire et l’unité de la Nation, pourquoi les porte drapeaux ne sont ils pas aidés financièrement par l’État pour incarner la mémoire nationale ? Par ailleurs, le ministère de l’intérieur ne pourrait il pas créer une section spéciale au sein de la réserve opérationnelle ou de la réserve civile, pour faciliter la participation aux commémorations et renforcer le lien entre le monde combattant et la communauté nationale ? Excellent ! La parole est à Mme la secrétaire

Tout d’abord, le ministère confie à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) le soin de contribuer au financement de l’acquisition et de la rénovation des drapeaux des associations d’anciens combattants. Après avoir été doublé en 2023, année au cours de laquelle le financement était passé de 150 à 300 euros pour une acquisition et de 80 à 160 euros pour une réfection, le montant de l’aide connaît une nouvelle évolution importante L’aide forfaitaire est remplacée par une aide proportionnelle aux dépenses engagées par l’association. Celle ci s’échelonnera désormais entre 100 et 500 euros.

L’ONaCVG propose aux associations et collectivités soucieuses de recruter de former des jeunes pour assurer le renouvellement des porte drapeaux. C’est dans cet esprit que les projets locaux de formation de porte drapeaux sont subventionnés et que, chaque année, à l’occasion du 14 juillet, est organisé un séjour

ont quitté le pays, mettant fin à plus de dix ans de lutte anti djihadiste de la France au Sahel. Lors d’une audition au Sénat en octobre dernier,

En effet, en plus des soldats, plus de 2 500 conteneurs auraient été évacués hors du pays. Une partie du matériel a rejoint la France par avion depuis la base de Niamey. Une autre partie a été transportée par la route, en passant par le Tchad jusqu’au port de Douala. Cette opération logistique aurait été assurée par un transporteur externe et civil. Une dernière partie, enfin, a été stockée dans la base militaire française de N’Djamena. Ce matériel devait être définitivement ramené dans l’Hexagone dans le courant du mois de janvier 2024, avec l’aide du Qatar.

Quel est le coût exact du désengagement militaire ? Enfin, quels sont les dispositifs prévus pour assurer la préservation des emprises françaises au Niger – ambassades, lycées ? Plus généralement, comment seront sécurisées les emprises françaises à l’étranger ?

La restitution de la dernière emprise militaire s’est déroulée dans les temps, le 22 décembre 2023. Vous interrogez le Gouvernement sur le coût de la manœuvre logistique de désengagement. Celui ci est de

démontables ou vétustes, de matériels logistiques, de stations d’épuration ou encore de bungalows et de structures de tentes, dont la valeur représente moins de 2 % du matériel français stationné au Niger.

Toutefois, la moitié des 1 500 personnes désengagées du Niger en deux mois par la route ou par les airs ont transité par le Tchad. Il s’agit donc d’une manœuvre, non pas de redéploiement, de transit. Vous soulevez la question de la sécurisation de l’ambassade de France. Les armées ont aidé au désengagement de l’ambassade, mené par la mission diplomatique de défense. Ainsi, 9 personnes, un conteneur et 9 véhicules ont été évacués par voie aérienne, civile et militaire, le 30 décembre dernier. La sécurité des emprises diplomatiques relève de la direction de la sécurité diplomatique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le ministère des armées a cependant renforcé le dispositif assuré par les gendarmes

comme l’augmentation régulière des besoins, une pyramide des âges très défavorable et des niveaux de rémunération et des perspectives d’évolution professionnelle peu attrayants.

découle de la transposition en droit français de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, laquelle s’impose à l’ensemble des États membres.

Par ailleurs, le système d’équivalences que vous citez, qui est défini à l’article L. 221 1 du code de la route et qui permet à certaines personnes de conduire des véhicules agricoles sans être

programmée le 15 avril prochain, l’absence de conformité de la gare maritime de Dzaoudzi aux normes internationales de sécurité ne risque t elle pas d’affecter le processus de reconduite à la frontière des étrangers à Mayotte ? Cette gare maritime est stratégique : elle a accueilli plus de 23 000 étrangers en situation irrégulière en 2023

Or, afin de loger les athlètes, ainsi que le personnel nécessaire lors des prochains jeux Olympiques et Paralympiques, le Gouvernement prévoit d’expulser près de 2 200 de ces étudiants. En guise de dédommagement, madame la ministre, vous leur avez promis 100 euros, ainsi que deux places pour assister à une épreuve olympique. Cette contrepartie est manifestement insuffisante, notamment pour couvrir les frais d’un éventuel déménagement.

Lors de la pandémie de covid 19, les étudiants et, plus généralement, les jeunes ont été les grands oubliés du Gouvernement, alors même qu’ils sont l’avenir de notre pays. Il me semble que vous délaissez de nouveau les étudiants, notamment les plus précaires, et que vous les sacrifiez à des fins publicitaires. Madame la ministre, le

L’auteur des faits, âgé de 18 ans à peine, est actuellement en détention provisoire. Le vendredi 15 mars, un autre jeune de 19 ans a été placé en détention pour vol avec violence.

travailler ensemble les professionnels de la sécurité, de la justice, du social et de l’éducation, afin d’élaborer le plan départemental de prévention de la délinquance. Ces assises se sont traduites par

d’une cartographie des dispositifs existants, l’élargissement de la démarche des cités éducatives, qui m’est chère, ou encore le renforcement de la formation des professionnels.

en décalage avec les annonces de votre gouvernement. La mobilisation d’ampleur pour un plan d’urgence pour l’éducation nationale en est une parfaite illustration. Cette situation rend d’autant plus cruciale la politique de la ville, dont les dotations sont en diminution, ce qui suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté balbynienne. Ainsi, alors que la population concernée par les prochains contrats de ville augmente de plus de 10 %, il n’est prévu aucun abondement supplémentaire du budget. Plus grave encore, le fonds qui permettait de soutenir financièrement les petites structures associatives en Seine Saint Denis, si précieuses, a été tout tout bonnement supprimé. Enfin, les élus et les responsables associatifs locaux constatent que la ville de Bobigny ne bénéficie, chaque année, que de 20 euros par habitant en quartier prioritaire de la

pour rétablir l’égalité républicaine entre toutes et tous. La citoyenneté, que votre gouvernement invoque sans cesse, mais qu’il réduit à de vagues incantations qui tendent à contrôler et réprimer toujours un peu plus les classes populaires, doit au contraire s’incarner par l’égalité républicaine. Aussi, quelles mesures comptez vous prendre pour renforcer les moyens de la politique de la ville en Seine Saint Denis, au regard de la forte hausse de la population destinataire et des besoins qui s’expriment ? Entendez vous poursuivre une véritable politique d’accompagnement des petites structures associatives, en remplacement du fonds d’initiatives associatives ? Enfin, renforcerez vous la dimension partenariale des contrats de ville

Le fonds d’initiatives associatives est un mécanisme qui permet également de soutenir les petites associations. Celui ci existe toujours et peut être mis en place s’il existe une volonté commune entre les services de l’État local et les collectivités. En ce qui concerne la question des moyens, je tiens à rappeler que, depuis 2020,

Mme Nathalie Goulet,

à ceux qui cherchent à diviser notre société et qui s’en prennent aux valeurs de la République, ainsi qu’à nos compatriotes juifs. Depuis plus de cinq ans, les gouvernements successifs luttent contre les islamistes, qu’ils soient liés à la mouvance des Frères musulmans

exige de la part des policiers que la poursuite d’un véhicule ne puisse être liée qu’à des faits d’une extrême gravité comme la fuite, l’évasion d’un individu dangereux la traque de l’auteur d’un crime de sang. Pour les autres situations, jugées moins graves, la course poursuite n’est pas obligatoire. Ainsi, avec l’aide de leur hiérarchie à travers la radio,

il est donc demandé à nos forces de l’ordre d’évaluer en quelques secondes la raison pour laquelle l’individu a refusé de s’arrêter, mais également l’éventuel danger d’une course poursuite

Par instruction de commandement en date du 14 mai 1999, la police nationale a rappelé que seules sont concernées les situations de fuite ou d’évasion d’un individu armé ayant l’intention d’attenter à la vie d’un tiers, de crime ou délits aggravés entraînant un préjudice corporel. Dans les autres situations pénales, toute poursuite systématique est exclue, notamment en cas de refus d’obtempérer. Cela se règle par une recherche ou une mise en surveillance de l’individu en vue de son interpellation. Depuis le 3 juillet 2020, cette doctrine d’intervention a évolué, et la préfecture de police autorise dorénavant la poursuite d’un véhicule refusant d’obtempérer. Cependant, cette poursuite s’effectue avec discernement et fait l’objet d’un compte rendu immédiat au centre interministériel de crise de l’intervention. L’instruction de commandement 89 vise spécifiquement, comme motifs de poursuite, des faits graves commis ou de nature à porter atteinte à la vie humaine ou à l’intégrité physique. Dans le contexte d’une poursuite de véhicule, l’avis hiérarchique est nécessaire, car les fonctionnaires de police doivent s’affranchir exceptionnellement du respect des règles du code de la route, dès lors qu’ils font usage de leurs avertisseurs dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Par ailleurs, des matériels récents et adaptés permettent de sécuriser l’action des policiers de terrain et d’apporter des preuves matérielles complémentaires à la justice. Le recours aux images de vidéoprotection en temps réel en est une illustration. J’espère, madame la sénatrice,

le maintien de l’offre de soins. En France, la voie d’accès à l’obtention du plein exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) est

envisagée pour faciliter le parcours de demande d’autorisation d’exercice de ces praticiens. Ces évolutions seront mises en œuvre pour partie à compter de la session 2024. En attendant, la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a permis une première réforme

Nous y sommes confrontés et cela entraîne déjà des défauts de soins. J’ai quitté mon officine ce matin avec près d’une quinzaine de patients diabétiques sans Trulicity et sans visibilité sur les

En 2021, un autre rapport appelait à réinvestir la santé mentale après le choc de la crise sanitaire. Les maladies mentales et troubles psychiques concerneraient 13 millions de Français, soit un sur cinq. Leur prise en charge est le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, devant celle des cancers, pour un coût annuel de 23 milliards d’euros. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime le coût économique et social des troubles psychiques à 109 milliards d’euros par an. Les rapports s’accumulent, les gouvernements se succèdent et la situation de la santé mentale en France ne fait qu’empirer, car les moyens, bien qu’importants, ne s’élèvent pas à la hauteur des besoins. Sur le terrain, cela se concrétise par des postes à pourvoir qui demeurent vacants, des fermetures de lits, des conditions de travail dégradées,

L’inventaire des maux ne permet pas de guérir, mais il témoigne de l’urgence à considérer la santé mentale comme une priorité gouvernementale. De surcroît, la carence de moyens ajoute au manque d’attractivité de la spécialité. Les professionnels de la psychiatrie considèrent que nous sommes assis sur des bombes à retardement entend il mettre en place à court et moyen termes pour attirer des personnels soignants et doter la santé mentale de moyens suffisants ?

inexorablement, quelque 70 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales sont décidés, fragilisant un peu plus l’équilibre financier du système de santé et du budget de la sécurité sociale. Cette situation accroît de fait la part de la prise en charge des complémentaires santé, et naturellement leurs tarifs, rendant aujourd’hui indispensables pour pouvoir se soigner. En effet, déremboursements par la sécurité sociale et hausses des primes des complémentaires vont de pair. C’est un véritable effet d’aubaine, dont certaines n’hésitent pas à profiter en pratiquant des augmentations hors de toute réalité. Ajoutons également l’impact non négligeable du niveau de taxation : 14,1 % pour les contrats solidaires, 21,1 % pour les contrats individuels. Cela contribue à alourdir encore un peu plus la note. Conséquence, les tarifs des mutuelles ont grimpé en ce début d’année +8,1 % et +10 % en moyenne ; +25 %, voire +30 % pour les catégories de personnes qui ne bénéficient pas de contrats collectifs, comme les retraités, les étudiants ou les indépendants. Cumulées à l’inflation et à la baisse du pouvoir d’achat, ces hausses de tarifs sont insupportables, faisant grandir le risque de non souscription à une complémentaire et, à terme, malheureusement, le risque de renonciation aux soins. Au niveau national, ce sont aujourd’hui 4 millions de personnes qui vivent sans complémentaire santé, 925 000 dans le seul département du Nord. Les récentes annonces du Gouvernement, comme le doublement des franchises médicales pour ne citer que cet exemple, tout comme l’explosion des dépassements d’honoraires chez certains praticiens, ne vont certainement pas arranger les choses. Madame la ministre déléguée, je reste convaincue que l’égal accès à la santé pour toutes et tous réside dans la prise en charge intégrale des soins par l’assurance maladie.

plusieurs dispositifs ont été mis en place par le Gouvernement. Je pense à la portabilité de la couverture santé pendant un an après la fin du contrat de travail ou encore la possibilité pour les branches de prévoir la prise en charge de tout ou partie de la couverture des anciens salariés.

que, pour les Français les plus modestes, nous avons mis en place la complémentaire santé solidaire (C2S). Grâce à elle, leurs dépenses de santé sont remboursées entièrement dans la limite des tarifs de la sécurité sociale.

Ce dispositif de coopération entre médecins généralistes et infirmiers a pour objectif d’améliorer la prise en charge de patients souffrant de pathologies chroniques. Il s’agit incontestablement d’une réussite, puisqu’il a permis de faciliter le parcours de soins du patient en valorisant de nouvelles compétences paramédicales tout en faisant gagner du temps aux médecins. C’est un magnifique exemple de délégation de tâches et cette réussite est reconnue de tous. La prise en charge des patients est excellente avec une écoute et une proximité beaucoup plus importantes, ce qui permet le dépistage plus précoce de certaines pathologies. Pourtant, la Caisse nationale de l’assurance maladie a acté la fin a acté la fin du financement des loyers pour l’hébergement des professionnels Asalée au 31 décembre 2023. Cette décision brutale, sans concertation, provoque un émoi important et une inquiétude légitime des professionnels mobilisés et des élus locaux. À cela s’ajoutent des situations surprenantes. Ainsi, dans la Nièvre, au mois de février 2024,

ces lacunes dans un rapport parlementaire. Deux ans après, de nombreuses victimes de la Dépakine, pourtant reconnues officiellement par l’Oniam, ne sont toujours pas indemnisées trente mois après cette reconnaissance. Pour une fois, ce n’est pas un problème de budget

afin de confier à un seul collège d’experts l’évaluation des responsabilités, de l’imputabilité et de l’étendue des dommages. Le nouveau collège a dû procéder, en plus de l’instruction des nouveaux dossiers, au réexamen d’un nombre important d’avis rendus précédemment. Ses travaux ont aussi été perturbés par la crise sanitaire.

témoigne de leur grande implication et a contribué à renforcer l’efficacité du dispositif. Ainsi, au 31 mars 2024, 1 946 victimes, dont 454 victimes directes, ont reçu une offre d’indemnisation pour un montant total de 85,8 millions d’euros.

Toutes les classes thérapeutiques sont touchées et ces pénuries en constante augmentation posent des questions quant à la garantie de notre sécurité sanitaire. La situation actuelle est non seulement aberrante pour les professionnels de santé sous pression, qui perdent du temps en recherches auprès des grossistes répartiteurs ou des confrères, mais elle est aussi, et surtout, dangereuse pour les patients, puisqu’elle menace à terme la prise en charge effective des personnes malades, avec un réel risque de perte de chances pour certains. Face à cette situation, une nouvelle feuille de route visant à garantir la disponibilité des médicaments a été présentée en février 2024. Mais l’augmentation constante de ces pénuries depuis 2017 suffit pour faire le bilan – sans effets ! – de ces plans à répétition. Je ne disconviens pas que la dernière en date présente un certain nombre d’actions susceptibles d’améliorer l’information et – je l’espère – d’apporter des solutions. Encore faut il qu’elles soient réellement appliquées ! Il faut notamment donner la possibilité aux pharmaciens d’officine de remplacer les médicaments en rupture par un médicament disponible sans solliciter le prescripteur sans solliciter le prescripteur qui est rarement joignable facilement. Il faut également assouplir les règles de fabrication à l’officine d’un certain nombre de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Les pharmaciens reçoivent une formation initiale et continue pour cela.

depuis 2019 en raison du contexte géopolitique et sanitaire international. Les ministres Catherine Vautrin, Frédéric Valletoux et Roland Lescure ont donc présenté en février dernier une nouvelle feuille de route destinée à lutter contre les pénuries de médicaments, qui fixe la stratégie gouvernementale des trois prochaines années.

dont l’article 24 accorde, au titre de la solidarité nationale, des trimestres supplémentaires pour la retraite des sapeurs pompiers volontaires ayant accompli au moins dix années de service. Cette disposition consacre une demande ancienne. Cette bonification de trimestres de retraite est tout d’abord une reconnaissance de la Nation pour l’engagement des sapeurs pompiers volontaires au service de la protection de la population. Elle permet aussi de renforcer l’attractivité du dispositif de fidélisation et de reconnaissance pour pérenniser la forme du volontariat et soutenir le recrutement. Cette mesure est surtout une mesure de justice sociale pour des citoyens qui acceptent pendant de nombreuses années des contraintes lourdes sur leur vie familiale et personnelle, parfois au péril de leur vie, se rendant disponibles plusieurs journées et nuits par mois, week end compris, pour porter secours à leurs concitoyens

du Gouvernement, qui entendrait réserver la bonification de trimestres aux sapeurs pompiers ayant des carrières hachées, ce qui écarterait la quasi totalité des sapeurs pompiers volontaires. Si cette orientation se confirmait, ce serait un détournement de la volonté exprimée sur toutes les travées du Sénat. Madame Madame la ministre, pouvez vous me confirmer que les bonifications de trimestres de retraite s’appliqueront à tous les sapeurs pompiers volontaires ayant effectué au moins dix ans de service et pouvez vous me donner la date à laquelle cette décision sera effective ? La parole

Le Gouvernement tiendra cet engagement, et ce de façon rétroactive : pour toute nouvelle liquidation de pension d’une personne ayant accompli par le passé au moins dix ans de service en tant que sapeur pompier volontaire, ces périodes donneront lieu à des trimestres supplémentaires, selon les conditions fixées par le décret.

La mesure permettra donc de corriger les interruptions de carrière et de garantir que l’engagement de ces volontaires ne pèse pas sur l’acquisition de droits à retraite. Cette avancée correspond bien à

engendrées par l’engagement en tant que sapeur pompier volontaire. Aller au delà de l’esprit du texte adopté à l’issue des débats relatifs à la réforme des retraites et accorder des bonifications de retraite aux sapeurs pompiers volontaires ayant des carrières

les projections pour 2024 laissent craindre un nouveau déficit de plus de 3 millions d’euros. Cette aggravation du déficit serait due, notamment, à une évolution des recettes de 1 %, qui est insuffisante pour couvrir l’inflation des dépenses. Par ailleurs, historiquement, il existe un sous financement de la psychiatrie en Charente. En effet, la Nouvelle Aquitaine y consacrerait en moyenne 175,10 euros par habitant de la région, mais seulement 146,20 euros par habitant en Charente. L’écart serait donc de 28,90 euros par habitant, soit un manque important pour le département en question, alors que les besoins en soins psychiques sont bien réels. Compte tenu des prélèvements à effectuer sur le fonds de roulement pour équilibrer le fonctionnement de l’établissement, le centre hospitalier Camille Claudel n’est plus en mesure aujourd’hui de réaliser son programme d’investissement qui a pour but d’humaniser ses locaux et de les rendre conformes à la réglementation. Pour toutes ces raisons, les instances dudit centre hospitalier demandent que la dotation annuelle annuelle de financement perçue soit, à tout le moins, mise au niveau de la moyenne régionale et qu’une aide à l’investissement d’ampleur soit attribuée pour répondre à la mise aux normes imposées

est de lui permettre de continuer à accueillir nos concitoyens touchés par des troubles psychiatriques dans des conditions d’accueil dignes et de qualité, en cohérence avec les orientations fixées par la feuille de route

a annoncé un déficit prévisionnel pour 2023, toutes activités confondues, de près de 1,15 million d’euros, cette projection ne tenait pas compte des crédits de fin de campagne 2023

Vous le savez, ces centres sont des structures de soins pivots et assurent une mission de service public. Depuis la fin des années 1980, l’association éducative du Mas Cavaillac, association d’utilité sociale intervenant auprès d’enfants, gérait l’antenne du centre du Vigan, et ce pour le secteur nord ouest du Gard comprenant Ganges et Saint Hippolyte du Fort. Depuis le début de l’été 2023, ce centre est fermé à la suite du départ du médecin psychiatre. Cette fermeture, qui était présentée comme temporaire, pose des difficultés de prise en charge pour la population ayant besoin de soins, évaluée à environ 500 enfants et adolescents. À ce jour, un médecin intervient de manière ponctuelle pour assurer la continuité du suivi des patients, mais aucun nouveau patient ne peut être accueilli. En effet, dans le Gard, le redécoupage de la psychiatrie est en cours d’arbitrage à l’ARS. Selon les nouvelles orientations, l’agence confierait la prise en charge de ce centre à l’hôpital d’Uzès, au détriment de l’association du Mas Cavaillac. Or aucun médecin d’Uzès n’accepte aujourd’hui de se rendre au Vigan, ni d’ailleurs à Ganges ou à Saint Hippolyte du Fort, faisant craindre la disparition définitive du centre.

tenu du nombre d’enfants concernés – près de 500 –, du bassin de population – 15 000 habitants –, de l’éloignement géographique du territoire, mais aussi de l’efficacité reconnue depuis près de quarante ans à cette association, je vous demande d’œuvrer à son maintien. La parole est à Mme la ministre

un complément de dotation annuelle de financement pour la gestion du CMPEA et, depuis 2022, elle sollicite l’État afin de bénéficier d’un complément de dotation pour conforter cette activité. Elle envisage même de reprendre les consultations au CMPEA de Saint Hippolyte du Fort, qu’elle gérait également jusqu’à sa fermeture en 2019. l’hypothèse privilégiée est plutôt de redonner la gestion du CMPEA au centre hospitalier d’Alès ou au centre hospitalier Le Mas Careiron. Une réunion s’est tenue en septembre 2023 avec la direction des deux établissements afin d’instruire la possibilité pour l’un des deux hôpitaux de reprendre le centre médico psychologique pour enfants et adolescents du Vigan. En attendant, une offre minimale est maintenue pour les situations les plus urgentes. En complément, il existe sur le territoire du Vigan un centre médico psychologique qui relève du centre hospitalier Mas Careiron et un hôpital de jour pour enfants géré par le centre hospitalier d’Alès. Une nouvelle réunion aura lieu au cours des prochaines semaines avec les élus du territoire et toutes les parties prenantes pour trouver les meilleures modalités d’organisation. Pour autant, je souhaite réaffirmer, au nom du ministre de la santé, qu’il n’est aucunement envisagé que l’activité du

et à proximité immédiate d’habitations résidentielles. Des actes de délinquance et des nuisances persistantes créent un contexte d’insécurité pour les enfants, le personnel éducatif municipal et les riverains du quartier. Cette situation réclame une attention toute particulière de la part du ministère. À la suite de différentes interventions de la municipalité, de la mobilisation des riverains et de la communauté éducative, l’État a annoncé le fléchage d’une enveloppe de 810 000 euros pour effectuer des travaux d’aménagement au sein de cette maison d’arrêt. Ils sont en cours. Plus globalement et à long terme, c’est la question de l’avenir de la maison d’arrêt qui se pose. Celle ci connaît une surpopulation préoccupante, avec 370 détenus pour une capacité de 180 places, soit un taux d’occupation de plus de 200 %. Le surpeuplement de la maison d’arrêt pose de réelles difficultés pour l’ensemble du personnel, engendrant de nombreux trafics et des problèmes de cohabitation caractérisés par des violences en tout genre. Au delà des travaux engagés et à poursuivre, ma question porte sur vos intentions pour traiter ce problème de surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de Béthune, dont on parle depuis des années, voire des dizaines d’années. moi apporter une réponse en matière d’infrastructures pénitentiaires pour répondre aux besoins du deuxième tribunal judiciaire des Hauts de France, qui touche plus de 600 000 habitants.

la construction d’un nouvel établissement sur la commune de Béthune n’est pas prévue. En revanche, trois nouveaux établissements sont programmés dans la région : à Saint Saulve, un établissement de 700 places ; une structure d’accompagnement vers la sortie de 120 120 places à Loos ; un établissement de 180 places à Arras. Vous pouvez compter sur la vigilance du garde des sceaux, madame la sénatrice, pour apporter les meilleures réponses à la situation carcérale de Béthune et de sa région. La parole

Ce centre souffre également, comme d’autres, d’un défaut d’encadrement, puisqu’il manquerait presque trente surveillants. Manque d’encadrement et surpopulation carcérale nourrissent des conflits, de la violence, tout en empêchant de mettre en place des programmes de réinsertion qui fonctionnent. La réduction de la surpopulation carcérale doit notamment passer par un travail de réinsertion, qui permet d’éviter la récidive, donc le retour en prison. Il est par conséquent essentiel d’améliorer ce volet, notamment l’accès à l’enseignement supérieur. Or une circulaire de 2009 interdit toujours l’usage des clés USB, qui sont des supports indispensables pour des travaux universitaires. La France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en juillet 2023, pour ce problème de surpopulation. Au mois de mars 2024, le comité des ministres du Conseil de l’Europe a fait part de sa profonde préoccupation face à l’aggravation de la situation. Mettre un terme à la surpopulation carcérale ne passe pas nécessairement par la construction de places de prison, puisque plus on construit, plus il y a de détenus. Le comité des ministres invite ainsi la France à s’attaquer aux causes profondes du phénomène, en évaluant de manière détaillée l’impact des dernières réformes

La prison est devenue la dernière réponse, en bout de liste, à toutes les défaillances complexes de la société. On y trouve ainsi beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Afin de mettre en conformité nos conditions de détention, le Gouvernement compte t il actualiser la circulaire de 2009 ? Envisagez vous un mécanisme national contraignant de régulation

Au 1 janvier 2024, dix neuf établissements ont été livrés. Cela représente 4 103 places nettes. Près de la moitié des établissements du programme seront opérationnels au cours de cette année. Le garde des sceaux a demandé à la direction de l’administration pénitentiaire d’accélérer les transferts d’accélérer les transferts des condamnés vers les établissements pour peine afin de limiter la surpopulation de nos maisons d’arrêt, tout en garantissant la réponse pénale. Le taux d’occupation de ces établissements est passé de 90 % en moyenne à près de 97 % en trois ans, avec l’utilisation de plus de 4 000 places

Nous avons appris en fin d’année 2023 que l’académie de Guadeloupe perdrait 107 postes d’enseignants à la rentrée 2024 : 52 postes en moins dans le premier degré et 55 dans le second degré. L’argument invoqué est celui de la chute du nombre d’élèves. Pourtant, l’académie manque déjà aujourd’hui cruellement de moyens de remplacement et d’enseignants spécialisés, comme elle manque d’ailleurs de psychologues, de compétences psychosociales d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED). Par ailleurs, une grande partie de la communauté scolaire de Guadeloupe vient de milieux sociaux marqués par la précarité. Cela se reflète dans les résultats des évaluations nationales réalisées par les élèves de sixième au mois de septembre dernier, qui classent la Guadeloupe à la trentième place sur 33 académies français et en mathématiques. Sans surprise, malheureusement, les six dernières places du classement national sont occupées par les académies ultramarines. Je dis « sans surprise », car les territoires ultramarins sont ceux qui concentrent le plus de difficultés. Ces évaluations nationales, plus qu’une photographie du niveau des élèves, sont en réalité une photographie des inégalités sociales. Il est donc incompréhensible de vouloir supprimer des postes d’enseignant dans ces territoires,

afin de rattraper le retard sur l’Hexagone ? Madame la ministre, la cote d’alerte est atteinte dans les écoles en outre mer. Il est urgent d’agir ! La parole est à Mme la ministre

sur une instruction interministérielle du 19 août 2022 concernant la stratégie de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes.

parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Rossignol, soyons très clairs : la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités n’a transmis aucune consigne aux ARS concernant un éventuel arrêt des financements des programmes en lien avec l’éducation à la sexualité,

des actions régionales contribuant à la lutte contre les addictions pour 2023 insiste sur l’intérêt de poursuivre le financement des programmes probants et des interventions prometteuses, avec renvoi à l’instruction interministérielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, publiée en août 2022. Plus globalement, certaines ARS engagent des réflexions afin

Comment habiller Pierre sans déshabiller Paul ? Comment maintenir des moyens constants pour nos festivals, qui risquent d’être les victimes collatérales d’un heureux événement, et éviter toute annulation de dernière minute ? Madame la ministre, nous manquons cruellement de visibilité. Ainsi, dans mon département, comme dans d’autres, nous ne disposons pas de référent « festival ». Or nous avons besoin d’un pilotage sur les décisions qui ont été ou qui seront prises. À trois mois des jeux Olympiques et Paralympiques, rien ne semble avoir été prévu annoncé. Comment accompagner nos festivals dans ces moments si délicats ? Comment maintenir une offre culturelle dans nos départements et aider tous nos festivals, sans exception, petits et grands, et surtout comment rassurer leurs organisateurs ? Madame la ministre, ne transformons pas l’année 2024,

de la concentration en alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les préparations pour les cosmétiques, l’aromathérapie, les compléments alimentaires et la pharmacie issues de productions comme la lavande, la mélisse, le thym, la menthe poivrée et bien d’autres.

de remplacement au désherbage chimique dont nous disposons actuellement ne sont pas viables économiquement, surtout pour les petites structures, et entraînent une très forte hausse des prix. Les producteurs réclament un investissement massif dans la recherche de moyens de lutte efficaces contre les mauvaises herbes et les alcaloïdes de leur caractère urgent et complexe, nécessitent des moyens financiers importants. Il faut agir vite, car, selon les producteurs, une vingtaine de plantes phares des PPAM pourraient ne plus être cultivées en France. Encore plus grave : le maraîchage est également concerné.

le caractère cancérigène et génotoxique de ces substances, que l’on peut trouver dans les miels, les tisanes et les compléments alimentaires. C’est la raison pour laquelle des mesures de gestion des risques ont été mises en place. Des teneurs maximales réglementaires ont été adoptées et publiées dès le mois de décembre 2020.

jusqu’à la stratosphère, ou, plus récemment, de l’ensemencement des nuages par l’iodure d’argent, comme cela est pratiqué en Gironde, où l’on compte 137 générateurs. Ces diffuseurs envoient dans l’atmosphère des milliards de particules d’iodure d’argent afin de saturer les nuages et de transformer la grêle en pluie ou de réduire la taille des grêlons. La fiche toxicologique de l’iodure d’argent met en évidence que, malgré le manque d’études sur ce sujet, « la pulvérisation d’aérosols d’iodure d’argent peut entraîner une contamination des sols et des milieux aquatiques, dont on ignore actuellement l’impact sur l’environnement ». Or l’iodure d’argent se bioaccumule, notamment dans les sols, comme l’a mis en avant le laboratoire Environnements et du rapport insistent aussi sur le fait qu’il n’existe pas de réglementation encadrant la pratique. Le Gouvernement déclarait en octobre 2018 qu’« il n’existe pas de démonstration robuste de l’efficacité de cette technique ». Il n’est donc pas possible d’en évaluer la pertinence économique, car les bénéfices ne sont pas assurés.

Madame la ministre, avez vous prévu d’engager une politique de recherche sur les dispositifs d’ensemencement par l’iodure d’argent afin de faire la lumière sur leurs effets sanitaires et météorologiques ? Par ailleurs, au nom du principe de précaution, avez vous prévu d’encadrer cette pratique en attendant les conclusions

Ce type de procédé soulève des questions qui nécessitent de conforter les premières évaluations effectuées par l’Organisation météorologique mondiale sur son efficacité et surtout sur son innocuité

en plus du plan Eau ; enfin, dans le cadre du plan France 2030 et en matière d’innovation, près de 1,8 milliard d’euros sont mobilisés pour accompagner l’agriculture, notamment pour permettre son adaptation au dérèglement climatique. Vous le voyez, nous choisissons plutôt la voie de l’adaptation

dans les sites Natura 2000. Depuis le 17 novembre 2023, les préfets ont pour mission de procéder sans délai au recensement des sites concernés. Une instruction technique appelle ainsi à une application couperet des interdictions, à une contractualisation obligatoire des mesures agroenvironnementales et climatiques, voire à une conversion en bio. Nous sommes assez loin de la démarche concertée et volontaire choisie par la France lors de la création du réseau Natura 2000. Dans les Alpes de Haute Provence, les agriculteurs concernés nous font pourtant part de leur volonté d’ouvrir des discussions pour trouver des solutions concertées et contractualisées, adaptées aux réalités locales. Dans le secteur de la lavande, déjà touché par des épisodes climatiques et épidémiques, confronté à une très forte concurrence et aidé par la puissance publique en conséquence, les lavandiculteurs du plateau de Valensole sont fortement touchés par ces restrictions, sur un périmètre de près de 15 000 hectares, sans qu’aucune concertation ni contrepartie soient envisagées. Les arboriculteurs du département dénombrent plusieurs vergers situés dans des zones classées dans les zones Natura 2000. Or il faut rappeler, mes chers collègues, que bien des progrès ont été réalisés depuis 1999, notamment dans la nature et l’usage des phytosanitaires employés. Par ailleurs, et nous avons tout lieu d’en être fiers, des investissements importants ont été réalisés sur ces exploitations pour économiser la ressource en eau, entre autres, grâce à des procédés respectueux de l’environnement.

Madame la ministre, nos lavandiculteurs et arboriculteurs encaissent un coup supplémentaire. Aussi, je demande que des concertations soient ouvertes pour évaluer au mieux la possibilité de contractualisations locales tenant compte des progrès réalisés et, si besoin, pour mettre en œuvre des mesures d’indemnisation

Vous l’avez dit, la gestion des sites Natura 2000 repose sur des mesures de protection de la faune et de la flore, adaptées aux situations locales, formalisées dans des contrats et des chartes. Rappelons quelques chiffres : le réseau français Natura 2000 comporte un peu plus de 1 750 sites terrestres et marins, représentant une surface terrestre de 7 millions d’hectares au total, soit environ 10 % de la surface agricole utile nationale.

Vous faites référence à une instruction concernant la mise en œuvre du décret du 28 novembre 2022 relatif à l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000, qui a été envoyée aux préfets.

Ensuite, à long terme, dans le cadre de la décentralisation de l’autorité de gestion des sites Natura 2000, l’État veillera à assurer une articulation avec les régions sur l’examen et l’évaluation des objectifs de ces sites. Vous l’avez compris, notre objectif est clair

Merci